Permettez-moi plutôt d'insister sur trois points : le premier a trait au soutien au mouvement sportif. Nous abordons une année de transition qui doit traduire une concrétisation de la nouvelle gouvernance du sport. Il est nécessaire d'activer tous ses rouages dans nos territoires, afin que la nouvelle instance soit pleinement opérationnelle lors des jeux Olympiques et Paralympiques que nous organiserons en 2024. Madame la ministre, je souhaite lever deux interrogations

Jusqu'à présent, vous avez efficacement mobilisé des marges de manoeuvre pour amortir l'effet de ces dépenses. Mais la commission des finances est formelle : cette stratégie ne pourra pas perdurer pour faire face aux 860 millions d'euros de financements complémentaires attendus jusqu'en 2025. jusqu'en 2025. Pouvez-vous malgré cela nous confirmer que ce besoin de financement sera sans conséquence sur le budget dédié au sport pour tous, comme le Président de la République s'y était engagé ? La seconde interrogation porte sur le cas spécifique de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD). La dotation à l'Agence est stable en 2020, ce qui ne correspond ni au dynamisme de ses dépenses ni à l'ambition du Gouvernement en matière d'éthique du sport. Il s'agit pourtant d'une attente forte de nos concitoyens. Nous devons nous montrer à la hauteur des enjeux de la lutte antidopage mondiale. Madame la ministre, pouvez-vous également nous confirmer que l'ensemble des dépenses afférentes au déménagement du laboratoire d'analyses seront bien prises en charge par l'État ? Mon attention a été portée sur un montant non compensé en 2020, représentant près de 8 % des ressources de l'Agence. Qu'en est-il ?

Ce dispositif est ambitieux, et tient une place importante dans le projet du Président de la République pour notre jeunesse. Pour preuve, il vous a même demandé, monsieur le secrétaire d'État, d'accélérer sa mise en oeuvre : il concernera ainsi 150 000 jeunes en 2021, Mais comment le montant de 1,2 milliard d'euros requis sera-t-il dégagé ? Je connais les inquiétudes de nombre de mes collègues, membres notamment de la commission de la défense, Ne sera-t-il pas prélevé également sur les crédits d'autres ministères ? Je terminerai mon intervention en évoquant le soutien à la vie associative. Nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 78 : le levier le levier de financement que constitue le Fonds pour le développement de la vie associative doit être renforcé. Il s'agit en effet de conforter le nouveau mécanisme qui doit succéder à la dotation d'action parlementaire, mais dont les montants sont inférieurs de moitié. Il s'agit aussi de répondre au climat d'incertitude qui ronge le mouvement associatif, alors que la générosité des Français a marqué le pas en 2018. Soutenons donc cette initiative, fruit d'un travail ancien, en particulier de Jacques-Bernard Magner, Pour conclure, j'approuve l'équilibre général que traduit le budget proposé pour 2020. Mes interrogations portent essentiellement sur la trajectoire ultérieure et la façon dont le Gouvernement honorera ses différents engagements. La loi de programmation budgétaire annoncée pour le printemps constituera, à ce titre, un rendez-vous important. C'est pourquoi, mes chers collègues, sur ma proposition, la commission des finances a émis un favorable sur les crédits de la mission

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le débat sur les crédits du ministère des sports se présente sous des auspices différents de l'année dernière.

La situation est aujourd'hui différente : la gouvernance territoriale de l'ANS a été définie dans la loi et l'année 2020 marquera le lancement des projets sportifs territoriaux qui sont attendus par les collectivités locales. Le budget se compose de deux programmes : le programme 219, « Sport », destiné à financer les actions du ministère et la part étatique de l'Agence, et le programme 350, consacré aux infrastructures des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Je m'étonne de cette mesure, compte tenu du fait que le rapport des tiers de confiance n'a pas été rendu public, et qu'elle semble donc anticiper la confirmation du transfert du corps aux fédérations. Toute déstabilisation des CTS à quelques mois des JO de Tokyo constituerait une initiative périlleuse. un mot sur l'avenir du ministère des sports, qui nous soucie toujours autant. Après la création de l'Agence, le rapprochement de son administration déconcentrée avec les rectorats et la fusion de son inspection générale avec celle de l'éducation nationale et de la recherche, on peut s'interroger sur les missions et les moyens dont dispose encore le ministère. Le comité interministériel du 4 novembre a renforcé une certaine confusion entre ce qui relève de la politique sportive, y compris au niveau interministériel, et la préparation d'un grand événement sportif international. La préparation des JO de 2024 suit son cours, et nous sommes heureux de constater que les moyens nécessaires ont été mobilisés. Un point de vigilance concerne cependant le Stade de France, dont l'avenir reste incertain et dont la modernisation doit être à la hauteur de l'événement olympique. La préparation de nos athlètes constitue laprincipale interrogation de ce débat budgétaire.

Alors que la préparation de nos athlètes doit constituer une priorité absolue, il ne faudrait pas que la mise à plat des structures constitue un obstacle sur la piste de nos performances. Même l'objectif de « jeux propres » est aujourd'hui fragilisé, compte tenu des contraintes imposées à l'AFLD. Le nombre des prélèvements est d'environ 8 000, alors qu'il dépasse les 12 000 dans des pays de taille comparable. Si le site de Saclay a été officiellement retenu pour accueillir le nouveau laboratoire, le budget ne comprend pas de crédits de paiement pour financer le déménagement.

En somme, nous souhaiterions que le Gouvernement développe, pour les athlètes de haut niveau et pour les pratiquants, la même ambition que celle dont il fait preuve pour les infrastructures olympiques. Dans cette perspective, la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis de sagesse sur les crédits de la mission.

Cette année, ce programme comprend une action supplémentaire. Je note avec intérêt cette démarche, qui permet d'identifier les 30 millions d'euros consacrés au service national universel. Notre assemblée devra toutefois être vigilante concernant l'exécution de ces crédits, afin de s'assurer qu'ils n'empiètent pas sur ceux qui sont alloués à d'autres postes de dépenses de ce programme. J'espère, monsieur secrétaire d'État, que nous disposerons d'informations précises et régulières sur la mise en oeuvre de ce dispositif et sa traduction budgétaire. nos questions sont nombreuses sur le SNU. Lors de votre audition, monsieur le secrétaire d'État, vous avez indiqué qu'entre 20 000 et 30 000 jeunes seront concernés en 2020. Avec un coût par jeune de 1 500 euros, le budget oscille entre 30 millions et 45 millions d'euros, soit une hausse de 50 %. Pouvez-vous aujourd'hui nous indiquer précisément où les financements supplémentaires seront trouvés si le nombre de volontaires dépasse les 20 000 ? S'agissant des capacités d'accueil du séjour de cohésion, le Gouvernement semble avoir déjà des difficultés pour loger 20 000 à 30 000 jeunes. Or une classe d'âge représente 750 000 à 800 000 jeunes. Faudra-t-il construire des infrastructures dédiées et spécifiques ? Les infrastructures existantes suffiront-elles ? Le taux d'encadrement est aussi très élevé, avec un adulte pour cinq jeunes. En 2020, il faudrait 4 500 encadrants pour 20 000 jeunes, et 150 000 pour 750 000 jeunes. Comment les recruter ? Comment les fidéliser ?

Le retour sur l'investissement social global du service civique représente près de deux fois l'engagement initial de l'État. Certes, le budget du service civique est en hausse, mais il connaît une nette inflexion : +2 %, contre +12 % l'an dernier et +14 % en 2018. Or le nombre de missions reste insuffisant par rapport au nombre de demandes, avec, dans certains cas, trois ou quatre demandes pour une seule mission. Cette rupture risque de casser la dynamique du service civique. Si tel était le cas, il serait très difficile et coûteux de la relancer. Enfin, la phase 3 du SNU prévoit un engagement volontaire de trois mois à un an. Mais une mission de service civique ne peut avoir une durée inférieure à six mois. Par ailleurs, pour qu'elle soit utile au jeune et à la structure qui l'accueille, les associations nous indiquent qu'une mission ne doit pas avoir une durée inférieure à huit mois. Former un jeune, le rendre opérationnel prend du temps. Or il faut que la structure d'accueil puisse également tirer un bénéfice de cette mission. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous garantir que la mise en place du SNU ne va pas conduire à une pression pour réduire la durée des missions du service civique et, donc, leur coût ? Comme vous pouvez le constater, mes chers collègues, de nombreuses questions restent en suspens. C'est pourquoi la commission de la culture, de l'éducation et de la communication a émis un avis de sagesse sur les crédits du programme 163. Mes chers 163. Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps de l'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.

Cela conforte l'idée que les politiques publiques mises en oeuvre dans ce cadre sont un enjeu majeur, notamment en perspective de la grande échéance attendue dans ces prochaines années, à savoir les Jeux de 2024, ou encore du large déploiement, en 2020, du service national universel. Concernant les programmes 219, « Sport », et 350, « Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 », le ministère disposera ainsi de plus de 710 millions d'euros, soit, à périmètre d'intervention constant, une hausse de 9,8 de 9,8 %, représentant un peu plus de 65 millions d'euros, ce qui est tout à fait substantiel. Ce budget- il faut le rappeler et le souligner avec force -sera le plus important depuis 2006. Certains nous feront peut-être remarquer que l'augmentation du seul programme « Sport », d'un peu plus de 35 % par rapport à 2019, est principalement liée à un changement de périmètre, les crédits de rémunération des conseillers techniques sportifs étant désormais budgétés sur la mission. Certes, et nous pouvons d'ailleurs nous réjouir de la confirmation du maintien de la totalité des CTS dans leur poste pour 2020. Voilà qui devrait rassurer les fédérations. Mais au-delà de cette évolution, l'augmentation du budget est bien réelle puisque, à périmètre constant- je le répète -, nous constatons une hausse de 9,8 %. Un autre sujet de satisfaction pour ce qui nous concerne est la traduction dans ce budget des priorités de la majorité présidentielle pour : d'une part, développer la pratique sportive en concrétisant la nouvelle gouvernance du sport autour de l'Agence nationale du sport, dont la déclinaison territoriale sera progressivement mise en place au cours de l'année 2020 ; et, d'autre part, pour assurer la bonne préparation des Jeux de 2024, en procédant à une montée en charge des dépenses relatives à leurs infrastructures. L'année 2020 constitue en effet une année charnière, marquée par l'engagement des premiers travaux. Je m'attarderai quelques instants sur le programme 350. Je salue sa montée en puissance, avec un budget en augmentation de 35 % en autorisations d'engagement et de 98 % en crédits de paiement, l'inscription inédite de crédits alloués à la dimension « héritage » des Jeux, destinés notamment à financer le futur laboratoire de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui a vocation à faire rayonner la France au-delà de 2024. Cette augmentation permettra également la mise en oeuvre de mesures nouvelles, au premier rang desquelles la revalorisation des primes aux médaillés olympiques et paralympiques à hauteur de 10 %, venant ainsi compenser la fin de l'exonération à l'impôt sur le revenu de ces primes. Je veux profiter de cette tribune pour saluer d'un même mouvement les 500 premières collectivités labellisées « Terres de Jeux ». Ces collectivités s'engagent dans l'aventure des Jeux avec leurs habitants ; parmi elles, figurent 17 communes ou intercommunalités iséroises. Ce mouvement de grande ampleur, qui va emmener tout le pays vers cette grande fête du sport, où la France sera au centre du monde, démarre très concrètement sur tout le territoire avec cette annonce de labellisation. Au-delà du budget du ministère des sports, au-delà des chiffres qui traduisent un engagement important, je souhaitais vivement saluer ces collectivités qui s'engagent pour ces Jeux. Ce salut que je viens d'adresser serait serait bien incomplet sans un hommage aux dirigeants et bénévoles des 180 000 associations sportives qui jouent un rôle essentiel auprès de notre jeunesse. Ces associations trouveront un soutien accru auprès de l'Agence pour promouvoir le développement des pratiques pour tous, partout et tout au long de la vie. L'objectif de 3 millions de pratiquants sportifs affiché par le Gouvernement est ambitieux ; les associations y prendront toute leur part. Concernant le programme « Jeunesse et vie associative », nous constatons une réelle dynamique des crédits, en augmentation de 8,4 %, ce qui s'explique principalement par le financement du service national universel. La majorité présidentielle a fait le choix d'investir, en faveur de la jeunesse, dans le déploiement du SNU. Quelque 20 000 jeunes seront concernés en 2020. Ces quinze jours durant lesquels tous ces jeunes vont en côtoyer d'autres venus d'horizons, de quartiers, de territoires différents ne vont pas d'un seul coup bouleverser la société. Il s'agit cependant d'un pari sur le moyen et le long terme. Cet outil de rassemblement de la jeunesse, ce tremplin pour un engagement, portera ses fruits de manière constructive dans les années à venir. Nous serons par ailleurs attentifs à ce que ce service national s'articule favorablement avec le service civique, dont l'objectif consiste à toucher 145 000 volontaires en 2020, avec une poursuite de la montée en charge vers l'objectif de 150 000 jeunes. C'est une autre manière d'engager la jeunesse au service du collectif dans la continuité continuité du service national universel. Le budget alloué à la jeunesse et à l'éducation populaire reste stable, à hauteur de 71,6 millions d'euros. Quant aux fonds attribués à la vie associative, ils bénéficient d'une hausse substantielle : les crédits alloués au développement de la vie associative augmentent de 18,7 %, ce qui permettra, notamment aux dirigeants associatifs, de bénéficier de droits complémentaires pour la formation. Je saluais tout à l'heure les bénévoles qui s'engagent au sein des associations sportives. Il nous faut également rendre hommage aux 13 millions de bénévoles qui s'investissent au profit des 21 millions d'adhérents du million et demi d'associations, tous tous types confondus, que compte notre pays. C'est une richesse, qui classe la France parmi les pays les mieux dotés du monde en la matière. Je souhaiterais conclure sur cette note d'optimisme, en rappelant l'importance de cette mission « Sport, jeunesse et vie associative ». Ce qui se joue quasi quotidiennement sur tous les terrains de sport, dans les gymnases, dans les maisons des associations, c'est tout simplement l'apprentissage de la citoyenneté au sein d'une cité ; c'est le maintien des liens et de la solidarité au sein d'un village. Notre majorité est attachée à ce million et demi d'associations, et nous sommes fiers de réaffirmer nos convictions

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le budget du sport, derrière une augmentation en trompe-l'oeil principalement allouée aux dépenses des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024- et d'ailleurs insuffisante pour cet objectif traduit une dégradation continue du sport français qui inquiète ses acteurs. Restera-t-il un ministère des sports dans quelques années, notamment après 2024 ? C'est la première question qu'on est en droit de se poser, non seulement en raison de la nouvelle suppression de 42 postes en son sein, mais aussi du fait de la menace, qui persiste, d'un détachement des CTS vers les fédérations sportives, tout cela dans un contexte où l'Agence nationale du sport prend de plus en plus la place du ministère.

aux collectivités, dont les finances sont déjà exsangues et qui gèrent pourtant 86 % des infrastructures sportives de notre pays. Tandis que nous faisons face à un vieillissement des équipements sportifs, 42 % d'entre eux ayant près de quarante ans, il est impensable que leur renouvellement repose intégralement sur nos collectivités. C'est pourtant bien ce à quoi les budgets successifs du sport risquent de conduire.

d'un côté, un sport de masse à qui l'on demande de faire toujours plus avec moins ; de l'autre, un monde sportif professionnel, en tout cas dans certaines disciplines, où l'argent est bel et bien présent, et même de plus en plus abondant du fait des paris sportifs ou des retransmissions audiovisuelles. La logique autant que la nécessaire solidarité nationale et le souci d'efficacité voudraient qu'une véritable péréquation ait lieu entre ces deux mondes pour faire en sorte que le premier continue de se développer et d'alimenter le second. Or, après que le Gouvernement a fait revoter l'Assemblée nationale sur le déplafonnement des taxes, il ne nous est pas même possible ici, au Sénat, d'aborder le sujet pourtant central qu'est celui du financement du sport. Les bénévoles, les élus et les adhérents des clubs sportifs français devraient donc accepter

Si les perspectives que votre budget trace pour le sport français inquiètent, la situation de la vie associative n'a malheureusement pas grand-chose à lui envier. Après la brutale suppression des emplois aidés, la politique fiscale injuste de votre gouvernement a enfoncé le clou : de la suppression de l'ISF à la hausse de la CSG, les dons des particuliers ont chuté drastiquement, d'au moins 20 % entre 2017 et 2018. En parallèle, le désengagement public se avec une nouvelle baisse, et pas des moindres, des crédits affectés à cette ligne budgétaire. Tout cela dans un contexte où les associations sont davantage sollicitées par les citoyens ou les collectivités, bien souvent d'ailleurs, pour assumer les missions de service public que l'État abandonne. À cet égard, la suppression de la réserve parlementaire, dont les crédits n'ont pas été intégralement transférés vers le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) conduit à une perte nette pour les associations, à hauteur de 27 millions d'euros.

le service civique concentre toujours la plus grande partie des crédits, sans que le dispositif puisse être réformé pour toucher véritablement son coeur de cible, que ne constituent pas les étudiants diplômés du supérieur à la recherche d'expériences à valoriser, ou pour qu'un véritable contrôle visant à débusquer le salariat déguisé soit mis en place. Enfin, le service national universel est censé favoriser

: +10,7 % en autorisations d'engagement et +11,6 % en crédits de paiement. Si l'on est tenté de se réjouir pour ce parent pauvre du budget de l'État, le constat est néanmoins à nuancer, car, tout comme l'année passée, cette augmentation des crédits

de cet événement sportif d'envergure, que nous attendons tous, et qui nous permettra de mettre en avant tant notre pays que notre culture du sport. Mais, pour développer la culture et la pratique du sport sur tout le territoire, il est indispensable de maintenir des financements importants hors jeux Olympiques.

Il faut rappeler que la pratique régulière du sport est primordiale en matière de santé et de bien-être. Elle l'est également en termes d'éducation : le sport est une formidable école de la vie. Il favorise et véhicule des valeurs essentielles dans notre République. Nous devons donc y allouer un budget adéquat pour une pratique du sport encouragée et facilitée à l'endroit de tous nos concitoyens et, surtout, sur tous les territoires. Je tiens d'ailleurs à souligner que beaucoup de grands champions ont commencé leur carrière dans de petits clubs. Dans ce cadre, la vie associative est primordiale. Notre groupe Les Indépendants s'était déjà inquiété l'an dernier de la dotation très insuffisante du Fonds pour le développement de la vie associative. Quand on connaît l'importance du tissu associatif pour la cohésion de notre pays, on ne peut qu'en appeler à un budget plus ambitieux. Je tiens à saluer la mise en oeuvre cette année- enfin ! -du compte d'engagement citoyen, qui permettra de faire le pont nécessaire avec la formation professionnelle. Mais, encore une fois, nous devons être attentifs à son financement. Les 11,5 millions d'euros pour l'année prochaine pourraient ne pas être à la hauteur des engagements pris.

C'est louable. Cette première année sera un test intéressant, afin de calibrer les financements pour les années suivantes. Je souhaite évoquer la création de l'Agence nationale du sport. Elle marque un tournant dans notre politique du sport, à la fois pour la pratique de haut niveau celle, plus classique, qui touche chacun d'entre nous. Ces pratiques doivent être encouragées. Concernant les moyens humains, l'inquiétude est toujours de mise à propos des conseillers techniques sportifs. Nous resterons attentifs à leur sort et à la pérennisation des postes. des postes. Je terminerai en évoquant le soutien indispensable aux fédérations. Certains sports sont dans une situation confortable, car ils disposent d'une tribune médiatique et d'une manne financière leur permettant d'appréhender l'avenir. Il y a un réel besoin de

de licenciés en plus des 18 millions de licenciés actuels. Malheureusement, c'est le moment qu'a choisi le Gouvernement pour annoncer la remise en cause de notre modèle sportif français. On peut faire mieux d'État, en le modernisant, mais on ne peut pas faire moins d'État. Une certitude demeure : les prises de position actuelles risquent de nous emmener vers la fin du modèle sportif de certaines fédérations. Nous savons que nous pouvons toiletter ce modèle décidé par le général de Gaulle en 1960 après les résultats décevants des jeux Olympiques, qui avait créé les directeurs techniques nationaux, les conseillers techniques d'État et lancé les lois de programme sur les équipements sportifs. Néanmoins, les missions des fédérations ont évolué au-delà de l'organisation du haut niveau. Il leur a été reconnu des missions d'intérêt général et de service public, consignées dans une convention pluriannuelle d'objectifs, qu'elles mènent dans des domaines variés, pour le compte d'autres politiques publiques ministérielles, que ce soient la santé, le tourisme, les affaires étrangères, le développement durable, la recherche, l'intérieur, l'éducation nationale, la ville, l'agriculture, sans que ces ministères les financent Les fédérations sportives et les bénévoles maintiennent une activité dans des zones fragiles, rurales comme urbaines, en luttant contre la désocialisation et la désertification. Il s'agit là de missions d'intérêt général auxquelles aucune structure privée ne saurait se substituer, tant ces opérations offrent un manque de perspectives et de rentabilité.

les crédits de l'ANS, qui finance le sport pour tous dans les territoires, restent stables, voire diminuent légèrement, alors que ceux qui sont affectés aux ouvrages olympiques s'envolent

Bien entendu, les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont un formidable challenge, qui impulse une véritable dynamique et ne saurait être atteint avec brio sans les efforts financiers qui l'accompagnent. Et nous saluons cet effort Cependant, un budget va bien au-delà des chiffres inscrits sur le papier. Il est avant tout la traduction d'une volonté politique permettant de rendre opérationnelles, sur tout le territoire, des ambitions empreintes d'une véritable grandeur. Afin d'y parvenir, il faut cesser de négliger- c'est le cas depuis bien trop longtemps maintenant - les associations, les infrastructures, la participation de tous et de tout le territoire. En effet, c'est grâce à eux que le succès sera au rendez-vous. Il est primordial de créer une politique du sport en adéquation avec la réalité du terrain. On le voit, le financement du sport pour tous n'est n'est absolument pas le bénéficiaire de cette hausse du budget, alors que la perspective des JO devrait être l'occasion d'un véritable rebond dans ce

Or, nous le savons, les moyens existent. Les trois taxes affectées connaissent une dynamique exceptionnelle. Elles permettront de récolter 420 millions d'euros, dont 146 millions d'euros seulement iront au sport, le reste revenant au budget général. fallu déplafonner ces taxes ou en relever le plafond. Nous aurions ainsi disposé des recettes suffisantes pour financer l'ensemble des sujets qui nous préoccupent, notamment les propositions qui contribuent à aider le mouvement sportif à se moderniser, à diversifier ses pratiques, à soutenir les collectivités locales dans leur effort de développement des équipements mis à la disposition des clubs et de leurs pratiquants et, ainsi, à façonner un contexte favorable pour atteindre l'objectif des 3 millions de pratiquants sportifs d'ici à 2024, si cher vos yeux.

législatif. Par ailleurs nous demandons un jaune budgétaire retraçant l'effort financier global de l'État dans le domaine du sport, ce qui offrirait une vision interministérielle et objective de l'action du Gouvernement en faveur du sport. En ce qui concerne la vie associative, les règles du jeu budgétaire nous contraignent fortement et ne nous laissent, pour ainsi dire, aucune marge de manoeuvre. Nous prenons au sport pour donner à la jeunesse, et nous prenons à la jeunesse pour donner au sport Cela ne mène pas bien loin quand nous connaissons les difficultés de part et d'autre : sport dans les territoires, vie associative dans le sport. De nombreux points soulevés dans le cadre de cette mission restent en suspens et doivent nous interroger sur la viabilité, l'efficacité et la pérennisation des moyens. Nous assistons, avec ce budget, à un véritable désengagement de l'État à l'endroit des associations,

de façon cohérente, en impliquant toutes les parties prenantes autour des priorités définies au niveau national comme à l'échelon local. Comment développer de nouveaux outils et une capacité à soutenir davantage l'emploi associatif, madame la ministre ?

Comment le Gouvernement envisage-t-il précisément de traiter cette question puisque, depuis le changement de système, nous n'avons pas retrouvé le niveau d'engagement financier qui prévalait du temps de la réserve parlementaire et des emplois aidés ?

J'en arrive au terme de mon intervention. Vous l'aurez compris, nous nous rangeons à l'avis de nos rapporteurs pour avis sur les crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » de ce projet de loi de finances. Bien sûr, nous saluons, avec les égards qu'ils méritent, les efforts consentis par le Gouvernement en faveur du sport de haut niveau dans la perspective des grands événements qui nous tiendront en haleine, mais nous n'oublions pas les territoires, qui, au terme de ce budget, pâtissent une fois encore du manque d'épaisseur de l'exercice. Et je réitère ma demande d'engagement de votre part, madame la ministre, concernant notre proposition relative à la taxe Buffet. En tout état de cause, et sur chacun des points de vigilance que je viens de pointer, nous ne manquerons pas d'exercer notre droit de regard, sans nous dispenser d'appeler à tel ou tel aménagement souhaitable, le cas échéant, dans un souci de cohérence et de cohésion.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la problématique principale posée par le programme 163, « Jeunesse et vie associative », réside dans son déficit de cohérence et dans la difficulté à saisir quelle est la véritable vision du Gouvernement en faveur de la jeunesse et de l'engagement citoyen. L'illustration la plus évidente de ce constat est l'absence d'articulation réelle entre le service national universel et le service civique, alors même que ces deux dispositifs ont comme point commun de vouloir renforcer la culture de l'engagement. Pire, l'expérimentation progressive de l'un semble freiner la montée en puissance de l'autre. En effet, le service civique, pourtant bien identifié et estimé par les 16-25 ans, qui se disent enthousiastes à son évocation, semble avoir atteint un plafond cette année, faute de crédits suffisants. À cet égard, le nombre et la durée des missions auraient été affectés, freinant ainsi cet « enthousiasme » et questionnant les structures d'accueil quant à l'avenir du service civique. Afin d'atteindre la cible des 150 000 jeunes, 30 millions d'euros supplémentaires seraient nécessaires par rapport à la loi de finances initiale pour 2019, soit 17 millions de crédits en sus de ce qui est actuellement budgété. Or ces 30 millions d'euros correspondent précisément au montant alloué au SNU, qui doit concerner quelque 20 000 volontaires en 2020. Monsieur le secrétaire d'État, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, pouvez-vous clarifier la position du Gouvernement sur le service civique et son devenir ? Entendez-vous revenir sur la grande ambition initialement attribuée à ce dispositif ? À titre personnel, j'appelle votre attention sur le fait que le déploiement de dispositifs d'affichage, tel que le SNU, se fait au détriment d'une logique d'insertion par l'engagement, qui, par essence, ne peut avoir d'effets que sur le temps long. C'est cette même logique qui prévaut entre le pass culture et l'éducation artistique et culturelle. Nous avons eu ce débat en commission de la culture hier. Parallèlement, il convient de noter que le budget dévolu au SNU sera supérieur de 5 millions d'euros à celui qui sert à financer les projets associatifs, alors que la France compte 12,7 millions de bénévoles, 23 millions d'adhérents, et que le milieu associatif représente 1,8 million d'emplois. Encore une fois, n'est-ce pas disproportionné, au moment où la dépense publique est limitée ?

Malheureusement, cette exigence ne paraît pas vraiment partagée par le Gouvernement, les crédits dédiés à l'éducation populaire constituant à peine plus de 10 % du budget du programme. Monsieur le secrétaire d'État, comptez-vous mettre en place une stratégie visant à redynamiser l'éducation populaire, comme le préconise le CESE, en investissant notamment

depuis plusieurs années, le sport demeure le parent pauvre du budget de l'État. Force est pourtant de constater que le financement du sport dans notre pays repose sur des ressources particulièrement dynamiques.

et nous connaissons toutes et tous la frénésie financière qui s'est emparée du sport-business. Celle-ci, hermétique à toutes les conjonctures économiques, connaît une croissance aussi constante que soutenue année après année. Quel contraste avec le vieillissement que subissent un grand nombre de nos infrastructures sportives au sein de nos territoires ! Quel contraste avec la baisse des moyens à laquelle se sont heurtées nos associations sportives locales du groupe du RDSE, à l'instar de nombre de nos collègues sur ces travées, appellent à un rééquilibrage de l'affectation du produit des taxes destinées au financement du sport, afin qu'il bénéficie plus largement au sport amateur. En effet, le dynamisme de ces ressources fiscales ne doit pas uniquement servir à abonder le budget général de l'État. La solidarité entre sport professionnel et sport amateur doit s'exprimer plus clairement en matière budgétaire. Nous pourrions le faire d'autant plus aisément que, compte tenu des ressources croissantes générées chaque année, ce soutien accru au sport dans les territoires pourrait être accordé sans pénaliser outre mesure le budget de l'État. Nous appelons de nos voeux ce rééquilibrage, car le projet de budget qui nous est proposé n'apporte aucune réponse nouvelle à cet égard. Si les crédits de la mission sont en hausse, c'est parce qu'ils traduisent le respect de nos engagements financiers dans le cadre des Jeux d'été de la XXXIIIOlympiade de l'ère moderne. À la lecture des chiffres figurant dans ce projet de loi de finances, certains pourraient même interpréter l'insuffisance des moyens alloués au sport amateur comme un effet d'éviction qui bénéficierait aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Nous le savons tous, il s'agit justement de l'écueil à éviter lorsque l'on organise de telles manifestations, à l'égard desquelles l'opinion publique n'est plus nécessairement aussi enthousiaste qu'auparavant. Un tel message serait désastreux, alors que nous attendons justement de ces Jeux qu'ils soient un moteur pour encourager la pratique sportive amateur dans notre pays. Le Gouvernement a fixé un objectif ambitieux de 3 millions de pratiquants supplémentaires. Pour ce faire, il faut doter plus généreusement nos territoires et les acteurs locaux du sport. Dans le cadre de sa réforme de la gouvernance du sport et de la création de l'Agence nationale du sport, l'exécutif attend du secteur privé qu'il participe plus largement au financement du sport. nous n'avons aucune certitude pour le moment sur un tel engagement futur. En revanche, le désengagement de l'État en matière sportive, lui, prend chaque jour forme beaucoup plus concrète. Nos inquiétudes demeurent vives sur notre capacité, dans les prochaines années, à mettre en oeuvre une véritable politique publique du sport en France. Et l'on en vient à penser que la prochaine dilution du ministère des sports des sports au sein du ministère de l'éducation nationale n'est pas forcément une fable, lorsque l'on constate le transfert des personnels des directions régionales de Ce transfert fait craindre un affaiblissement des missions précédemment exercées par ces agents et un redéploiement de ces derniers au bénéfice du service national universel un SNU appelé de ses voeux par le Président de la République et qui bénéficie d'une attention particulière de la part de l'exécutif. J'en viens aux crédits dévolus au programme « Jeunesse et vie associative ». Nous avons pris connaissance des nouveaux moyens mobilisés pour la montée en puissance du SNU. Nous souhaitons toutefois rappeler notre attachement au dispositif du service civique, dont la pertinence ne fait l'objet d'aucune contestation. Le ralentissement très significatif des financements dédiés à ce dispositif nous fait craindre une réduction de la durée des missions afin de pouvoir toujours répondre à un nombre important de demandes. Nous rappelons que le déploiement du SNU ne doit pas pénaliser outre mesure la poursuite de la mise en oeuvre du service civique avec l'ambition qui a été la sienne jusqu'ici. De nombreuses zones d'ombre continuent d'ailleurs d'entourer l'avenir de ce dispositif. Nous attendons des éléments de réponse concernant la mobilisation et la répartition des places d'accueil, ou encore sur la question de l'encadrement et de la formation des encadrants. Au regard des lourds moyens financiers que le SNU devrait mobiliser dans l'avenir, sa redondance avec de nombreux dispositifs existants est en outre souvent pointée du doigt. Au-delà de ces griefs, nous sommes conscients du fait que ce projet de loi de finances, même s'il n'est pas porteur de ressources nouvelles pour le développement du sport dans nos territoires, a au moins le mérite de stopper l'hémorragie observée ces deux dernières années dans ce domaine. Il est également porteur du respect de nos engagements financiers en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Aussi, compte tenu de ces éléments, le groupe du RDSE s'abstiendra sur le vote

notre politique sportive se doit d'être un vecteur d'émancipation, de valeurs, de lien social. Nous restons convaincus que le sport de masse, la démocratisation du sport sont compatibles avec l'excellence, l'élite, le professionnalisme,

il est difficile de le comparer aux budgets des années précédentes. Des modifications fortes sont venues affecter la politique sportive : financement par le programme 219 des conseillers techniques sportifs, sans pour autant que le budget soit accolé à celui des personnels déconcentrés et de la direction des sports, ce qui manque de cohérence et affaiblit le ministère.

Un constat : à périmètre constant, les crédits du programme 219, « Sport », ont baissé de 11 % entre 2017 et 2020. Il est donc de notre responsabilité de mettre en adéquation les engagements affichés et les moyens pour les atteindre. C'est d'ailleurs ce que le Sénat a fait ce week-end, en adoptant, Claude Kern l'a rappelé, un amendement cosigné par des dizaines d'entre nous visant à accorder plus de moyens à l'Agence nationale du sport.

de 2024 ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. Il est nécessaire d'investir massivement dans la politique sportive pour tous et pour tous les territoires. C'est là que nous connaissons un véritable manque Sur ce point, nous avons quelques inquiétudes quant aux moyens donnés à l'Agence nationale du sport, qui, avec 284 millions d'euros en 2020, devra notamment se confronter aux objectifs affichés des fédérations sportives en matière de projets de performances ; l'enveloppe risque d'être insuffisante.

Par ailleurs, le financement du fonctionnement de l'ANS lui-même n'est pas précisément défini. Cela est dommageable, quand cette agence doit monter en puissance dans les prochains mois. Madame la ministre, l'Agence nationale du sport est un nouvel outil qui, j'en suis sûr, prouvera son efficacité. Ce n'est toutefois pas le seul sujet de notre discussion budgétaire. En effet, la politique sportive de l'État, vous nous l'avez rappelé, c'est aussi la politique sportive en direction de tous les citoyens, de l'école à l'Ehpad, de l'université à l'entreprise en passant par le monde médical. C'est également la politique sportive pour tous les territoires, en métropole comme outre-mer.

Je pense notamment au dispositif permettant aux entreprises de ne pas risquer de voir requalifier en avantage en nature leur engagement pour la pratique sportive. Pour les entreprises, la loi est plus sécurisante qu'une circulaire. aux différents dispositifs ambitieux visant à favoriser le mécénat à destination du mouvement sportif et des sportifs. Je pense enfin aux propositions pour une meilleure pratique du sport à l'école ou pour l'expérimentation de la prise en charge partielle des activités physiques prescrites par ordonnance.

Permettez-moi de penser que c'est aussi cela qui a conduit les commissions du Sénat à émettre un avis favorable sur le projet de budget qui vous est présenté aujourd'hui. L'historique récent du budget de mon ministère

Une telle politique pour la jeunesse et la vie associative nécessite, par nature, une mobilisation interministérielle. Là est la difficulté, si je puis dire, de cette discussion budgétaire : les crédits prévus dans cette mission ne constituent qu'une fraction des moyens qui permettent de mettre en oeuvre la politique en faveur de la jeunesse et de la vie associative. représente un investissement de 95 milliards d'euros. L'effort de l'État en faveur des associations, hors dépenses fiscales, s'élève à plus de 7 milliards d'euros. Cela devrait vous rassurer, madame

n'est pas le cas ! Cette politique revêt également une dimension partenariale forte. Sa construction s'appuie sur un dialogue soutenu avec les collectivités territoriales, d'une part, et les associations et fondations, d'autre part. Le programme 163 ne retrace donc qu'une fraction de l'effort de la Nation dans ces domaines, mais il permet à l'État de jouer un rôle essentiel d'impulsion et d'innovation, de professionnalisation, de coordination interministérielle, d'expertise et de régulation. Dans ce programme, quatre séries de mesures pour la jeunesse méritent d'être mises en avant. La première porte sur l'accès à l'information, avec, notamment, le déploiement de la nouvelle « boussole des jeunes ». La deuxième concerne la mobilité internationale, levier important de l'intégration sociale et professionnelle et de l'émancipation des jeunes. Dans ce domaine, nous renforçons la lisibilité de nos dispositifs et leur accessibilité pour les jeunes. La troisième a trait au développement des accueils collectifs de mineurs et des accueils de loisirs, qui permettent l'ouverture culturelle, sportive, et favorise l'inclusion sociale. Ce sont 108 millions d'euros par an qui seront investis pour soutenir les collectivités dans la mise en oeuvre du plan Mercredi. Enfin, il m'est impossible de parler de la jeunesse sans évoquer le service civique et le service national universel. Le service civique représente une formidable école de la vie, de l'engagement, qui attire chaque année plus de jeunes.

Les associations occupent une place essentielle dans la vie collective de la Nation et le fonctionnement de notre modèle de société. Avec 21 millions d'adhérents, 13 millions de bénévoles, mais aussi 1,8 million de salariés, soit près de 10 des emplois, ce secteur est, à la fois, un ferment de cohésion sociale et un acteur économique majeur. Les associations sont au coeur du projet de société de l'engagement porté par le Président de la République. C'est un nouvel

Depuis lors, les personnels pédagogiques et techniques qui continuent à relever de l'État sont rémunérés par lui, alors que la rémunération des agents titulaires en Creps ayant opté pour l'intégration ou le détachement dans la fonction publique territoriale au 1 janvier 2020 doit être compensée par l'État aux régions, puisque ce sont elles qui paient désormais ces personnels. Entre 2017 et 2020, plus de 12 millions d'euros ont été progressivement intégrés de manière pérenne dans les dotations générales de fonctionnement versées aux régions.

dans certains territoires, mais que cette régionalisation contribue à accroître les inégalités dans un certain nombre de domaines. J'y suis d'autant plus sensible que je vis dans une région,

Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.